à l'enseignement primaire, une volonté constante et réaffirmée de notre assemblée : nous considérons qu'oeuvrer en faveur de l'enseignement primaire est une priorité absolue. Ce soutien se traduit par une

mais une absence de couverture géographique risque de poser le problème de l'égalité des territoires. La troisième raison pour laquelle nous soutenons votre budget est spectaculaire

en sixième, ce qui est intéressant. Elle atteint 44 % en éducation prioritaire, ce qui révèle une prise de conscience de la nécessité de s'appuyer sur l'école pour rattraper un éventuel retard.

le temps s'égrène inexorablement. Au service de cette politique, vous avez pris des mesures financières pour les revenus des enseignants. Je vous en félicite, car, autant le dispositif

Je souhaite également attirer votre attention sur le nombre insuffisant d'enseignants référents, chargés de mettre en oeuvre et de faire vivre les projets personnalisés de scolarisation. Ces projets doivent être une réalité pour tous les élèves en situation de handicap, y compris ceux qui ne sont pas accompagnés par un AESH.

Ces suppressions ont été compensées par des heures supplémentaires. Or le recours aux heures supplémentaires entre dans une phase très tendue, car nous sommes dans le pic démographique des enfants de la décennie 2000, désormais au collège et au lycée. Il faut s'intéresser aux difficultés singulières de chaque établissement. Entre les enseignants à temps partiel et ceux dont l'état de santé ne leur permet pas de faire des heures supplémentaires, l'enveloppe des heures supplémentaires annualisées (HSA) porte souvent sur une petite moitié des enseignants de chaque discipline. En raison de cette concentration, il n'est pas rare qu'un chef d'établissement demande à un enseignant d'effectuer trois, voire quatre heures supplémentaires hebdomadaires. Le vivier sur lequel s'appuyer se réduit de plus en plus.

y êtes attaché. Les professeurs ne sont pas assez formés à cette mission. Leurs formations initiale et continue doivent être renforcées et améliorées. La transmission des valeurs républicaines engage collectivement et à long terme chaque établissement. À cet égard, la journée de la laïcité, le 9 décembre, doit être un temps fort d'unité dans nos établissements scolaires. L'enseignement de ces valeurs doit fédérer les équipes pédagogiques et l'ensemble des disciplines.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'excellence de l'enseignement agricole et sa capacité d'insertion sociale et professionnelle sont reconnues par tous. technique agricole », ne sont pas à la hauteur des défis que doit relever l'agriculture. Je pense à la nécessité de renforcer la résilience et la sécurité alimentaire, à la volonté de produire et transformer autrement.

agricole, qui connaissait un lent déclin depuis quelques années, s'est brutalement dégradée cette année. De fait, il a été très fortement touché par la crise financière et économique de la covid-19 : les pertes sont estimées à plus de 45 millions d'euros

Il est de plus en plus concurrencé par des formations de l'éducation nationale, tandis que la pression sur les équivalents temps plein (ETP) empêche tout dynamisme : pour ouvrir une nouvelle filière dans un établissement, il faut aujourd'hui en fermer une autre.

Autre conséquence directe des restrictions financières et humaines : la réforme du baccalauréat ne peut pas se déployer dans de bonnes conditions. Par manque de dotations horaires, les chefs d'établissement ne peuvent proposer qu'une doublette de spécialités en terminale ceux qui font le choix de proposer deux doublettes le font au détriment des options proposées. Cette situation est inacceptable : il y a rupture d'égalité de traitement entre lycéens Enfin, le budget 2021 ne répond pas aux problèmes que nous signalons depuis plusieurs années : la revalorisation des agents de catégorie 3 et le différentiel de traitement des assistants d'éducation.

L'enseignement agricole est donc l'un des rares secteurs ayant perdu des crédits en 2020. Pour toutes ces raisons et pour tirer vigoureusement la sonnette d'alarme, la commission de la culture a émis, de façon unanime, un avis défavorable sur les crédits du programme 143.

prend bien peu en compte la crise sanitaire qui se prolonge en une crise économique et sociale très profonde. En termes de moyens humains, par exemple, rappelons que les 2 039 postes supplémentaires budgétés pour le premier degré sont pour la plupart, comme il vient d'être rappelé, issus de la mobilisation du Sénat pour qu'aucune classe ne ferme en milieu rural sans l'accord du maire. Souvenons-nous aussi des batailles menées par certains d'entre nous pour empêcher des fermetures de classe décidées en plein confinement, au moment même où tout le monde s'inquiétait des possibles décrochages à venir. de postes demeurent insuffisantes, y compris au regard de vos propres objectifs. Par ailleurs, elles sont à mettre en parallèle avec la suppression de 900 postes de stagiaire. Enfin, elles se font détriment du secondaire, où 1 800 postes sont supprimés, en contradiction avec la réalité démographique et la nécessité d'un accompagnement renforcé pour faire face aux réformes qui bousculent profondément, en particulier, Au motif de compenser ces suppressions, vous industrialisez les heures supplémentaires, qui atteignent près de 10 % du temps d'enseignement ! Si, sur le papier, vu du ministère, cet allongement du temps de travail des enseignants semble fonctionner, la réalité est tout autre plus de 12 millions de crédits d'heures n'ont pas été consommés en 2019, et des expériences toutes plus kafkaïennes les unes que les autres nous remontent des établissements, qui ne parviennent pas à les réaliser concrètement.

Aux moyens nécessaires en termes d'enseignants je pourrais ajouter le soutien aux directeurs d'école, qui n'est pas du tout à la mesure des tâches qu'ils ont à réaliser dans le contexte actuel, ni des SOS qu'ils ont lancés avec force ces derniers temps- tout cela malgré vos annonces.

pour l'inclusion scolaire) ne sont toujours pas comptabilisés dans les effectifs généraux dans toutes les académies. C'est inhumain au sens propre du terme ! C'est aussi profondément injuste, car cela ôte des moyens aux établissements, alors qu'il leur en faudrait, au contraire, davantage. J'en viens au plan de revalorisation des enseignants, qui n'est absolument pas de nature à répondre à la crise de recrutement que nous traversons. Ainsi, alors qu'un professeur certifié, dont le dont le temps de travail est estimé à 44 heures hebdomadaires, est payé environ 1 600 euros, croyez-vous réellement qu'une revalorisation qui va se résumer, pour les deux tiers des enseignants à une prime informatique de 150 euros par an va susciter de nouvelles vocations ? Par ailleurs, pourquoi vous obstinez-vous à refuser de piocher dans les listes complémentaires aux concours pour faire face aux postes non pourvus dans certaines disciplines ou académies ? Nous disposons là de personnels motivés et disponibles, qui ont déjà un pied dans la formation ! Monsieur le ministre, je suis un peu stupéfaite que vous ayez choisi de faire des annonces très inquiétantes sur l'éducation prioritaire au moment où plus d'une centaine de maires, dans une très large diversité politique, alertent sur les risques de décrochage de certains de nos quartiers et sur la nécessité que le plan de relance accorde une attention toute particulière à ces quartiers- et plus qu'une attention : des moyens. Oui, il y a besoin de remettre le chantier de l'éducation prioritaire sur la table, car trop de communes, d'élèves et de familles qui devraient en relever en sont exclus. Non, les difficultés sociales ne sont pas l'apanage des milieux urbains, mais ce chantier doit être guidé par la promesse républicaine d'égalité et l'affirmation de notre République sociale. Car défendre la République, c'est aussi refuser une République à la carte, où tout se contractualise et se négocie dans une concurrence d'autant plus redoutable qu'elle vise à se partager des moyens qui manquent. Je terminerai en abordant la situation des collectivités territoriales. Les 100 millions d'euros qui leur sont affectés vont essentiellement répondre à l'instruction obligatoire à 3 ans et à son corollaire de compensations

La nécessaire mobilisation de la société autour de son école se manifeste dans le budget de l'État, dont elle constitue le premier poste de dépenses. Plus récemment, elle s'est également traduite par des mesures que nous soutenons l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans, l'obligation de formation des jeunes jusqu'à 18 ans et, bien sûr, le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+. Sans oublier un socle élargi et affermi, que vous avez baptisé, monsieur le ministre, l'école de la confiance. Un socle élargi et affermi, mais un socle perfectible. Je pense à l'éternel problème du zonage des REP et REP+ : certaines écoles, dites orphelines, en sont exclues, surtout en zone rurale, alors qu'elles devraient pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique. Dans ces conditions, nous serons très attentifs à l'expérimentation de la suppression de la carte REP. Si l'idée est de rebattre les cartes pour coller au mieux aux besoins réels des établissements, nous ne pourrons que la soutenir. soutenir. Le socle de l'école de la confiance est aujourd'hui mis à mal par la situation sanitaire. C'est bien ce qu'ont prouvé les évaluations de cette année en CP et CE1 : elles ont mis en évidence un creusement de l'écart entre les élèves en éducation prioritaire et les autres. Le confinement a donc eu pour ces derniers un effet négatif ; il a, en quelque sorte, annulé les effets bénéfiques du dédoublement des classes. La leçon est sans équivoque : si l'école de la République peut compenser un environnement sociologique défavorable, c'est à la condition qu'elle soit physiquement présente. Ce qui ne signifie évidemment pas qu'il faille manquer le virage de l'école numérique. La création d'une dotation informatique de 150 euros par enseignant prouve d'ailleurs que le Gouvernement en a bien conscience. Certes, 150 euros, cela peut paraître peu, mais le montant importe moins que le signal envoyé : celui d'une mutation du métier d'enseignant et de l'école tout entière. Les grandes orientations tracées pour cette école de la confiance nous semblent donc aller dans le bon sens, à condition de ne pas négliger le secondaire. Nous comprenons bien que la priorité soit donnée au primaire, mais cela ne doit pas nous faire oublier que le niveau des élèves ne s'apprécie pas uniquement au travers du français et les mathématiques. En tant que présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes, j'aimerais mettre l'accent sur une problématique spécifique au secondaire les cours d'éducation sexuelle. Le code de l'éducation prévoit que les élèves doivent avoir trois rendez-vous sur ce thème au cours de leur scolarité. Monsieur le ministre, est-ce effectivement le cas ? La loi sur les cours d'éducation sexuelle est-elle respectée sur tout le territoire de la République ?

En miroir de l'école de la confiance se construit aussi une école de l'inclusion, ce qui soulève toute la problématique des AESH. Plus de postes, c'est bien, mais une approche du sujet exclusivement quantitative n'est pas satisfaisante. D'un point de vue qualitatif, il faut se poser la question de la formation et de l'attractivité du métier. la qualification, nous ne pouvons que saluer la mise en place d'une véritable formation, mais celle-ci demeure incomplète. Par exemple, les AESH ne sont pas formés, ou peu, aux enfants atteints de surdité. concerne l'attractivité, il faut rappeler que la rémunération des AESH est très faible, de l'ordre de 600 à 800 euros par mois. À cet égard, gare aux fausses bonnes idées on ne rendra pas plus attractif ce métier en encourageant les AESH à accompagner plusieurs enfants en même temps, sans prendre en compte les difficultés de mobilité. L'école de l'inclusion est donc encore perfectible. Je terminerai en évoquant l'enseignement technique agricole. Que dire, si ce n'est que le constat est amer ? L'enseignement technique agricole ne représente que 2 % des crédits de la mission « Enseignement scolaire ». Amer, le constat l'est d'autant plus que le gouvernement auquel vous appartenez n'a eu de cesse de valoriser les agriculteurs, leur fonction nourricière de la Nation et leur rôle déterminant dans la crise sanitaire que nous traversons. Or la crise de la covid a particulièrement affecté l'enseignement agricole et pose désormais la question de sa survie. Menaces de fermetures de classe, impossibilité d'ouvrir de nouvelles filières sans en fermer d'autres,

Force est de constater que les élèves de l'enseignement agricole sont les laissés-pour-compte de ce budget. Ils représentent pourtant l'avenir de l'agriculture ; à ce titre, pouvoir être formés aux nouveaux enjeux technologiques et environnementaux, afin que notre agriculture reste l'une des meilleures du monde. Comme l'a souligné la rapporteure pour avis, Nathalie Delattre, que je salue pour la qualité de son travail, tous les arbitrages en faveur de l'enseignement agricole ont été perdus au bénéfice de l'enseignement général. Eh oui ! De surcroît, un déséquilibre persiste entre les enseignements agricoles public et privé : alors même que ce dernier accueille plus d'élèves, il reçoit

Ce choix est d'autant plus regrettable qu'il intervient au moment où l'État lance « 1 jeune, 1 solution ». Quelle sera la solution pour les jeunes dans l'enseignement technique agricole ? ? La situation est telle que la survie de l'enseignement agricole est, semble-t-il, en jeu. C'est pourquoi, monsieur le ministre, si le groupe Union Centriste

Monier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est dans un contexte bien compliqué pour l'éducation nationale que nous étudions la mission « Enseignement scolaire L'assassinat de Samuel Paty, l'un des siens, a profondément ébranlé la communauté enseignante, dont les membres ont été meurtris dans leur chair. Je crois que nous n'avons pas encore suffisamment pris la mesure, collectivement, de ce que cela a représenté pour eux. Les hussards noirs de la République sont les piliers de notre société face à l'obscurantisme. Ils ne manquent ni de courage, ni de volonté, ni de conviction pour remplir cette mission. Il faut entendre leurs alertes lorsqu'ils disent ne pas se sentir assez protégés ni soutenus et avoir besoin de davantage de formations pour répondre sereinement aux nombreuses questions de leurs élèves. Cette violence s'ajoute à un contexte difficile pour les personnels de l'éducation nationale, en première ligne dans cette crise sanitaire et aux prises avec des situations complexes à gérer des protocoles difficiles à mettre en place et communiqués tardivement, un stress important, des élèves en difficulté après le confinement, et des parents inquiets. Et ce alors que les obstacles dans un contexte ordinaire sont nombreux classes surchargées, réformes difficiles à mettre en oeuvre, manque de matériel, et un sentiment profond que leur travail n'est pas reconnu. Les directeurs et directrices d'école étaient déjà à bout avant la crise sanitaire car leurs missions sont trop nombreuses. Nous n'avons pas oublié la mort de Christine Renon lors de l'année scolaire précédente ni les mots bouleversants qu'elle nous a laissés. Il n'est pas question qu'un tel drame se reproduise. Tendez l'oreille, monsieur le ministre ! Entendez-vous la souffrance des enseignantes et des enseignants ? Notre école de la République a pour mission de fournir à nos élèves un enseignement qui permette de résorber les inégalités. Or elle n'y parvient plus, malgré la bonne volonté de celles et ceux qui la font vivre. La plus belle de nos institutions souffre

hausse n'est pas significative, car elle correspond au transfert d'une partie du budget consacré au sport et à la jeunesse ainsi qu'à une revalorisation salariale. Nous nous interrogeons d'ailleurs sur cette revalorisation, certes positive, mais qui ne concernera pas tout le monde et sera dégressive. Nous regrettons que vous n'ayez pas plutôt fait le choix d'augmenter le point d'indice pour tout le monde. Quant à la prime d'équipement, l'objectif annoncé est de permettre le renouvellement d'un équipement informatique complet. 450 euros sur trois ans, est insuffisante pour y parvenir. Les crédits alloués à la mission « Enseignement scolaire » prévoient une hausse du nombre de postes d'enseignants dans le primaire, notamment afin de poursuivre le dédoublement des classes dans

Ces créations de postes en primaire sont une bonne chose, mais malheureusement, force est de constater que cela se fait au détriment du dispositif « Plus de maîtres que de classes », qui bénéficiait notamment aux écoles rurales, et que ces créations entraînent des suppressions de postes ailleurs. Ce budget prévoit aussi de mettre en place des décharges pour les directeurs et directrices d'école. Est-ce un effort suffisant pour répondre aux besoins réels ? Nous en doutons.

complexe des réformes des lycées général et professionnel. Monsieur le ministre, vous nous avez expliqué que ces suppressions sont compensées par le recours aux heures supplémentaires. Mais les enseignants comme les chefs d'établissement alertent sur le fait qu'ils ne sont pas en capacité d'absorber autant d'heures supplémentaires. D'ailleurs, une grande partie des heures supplémentaires actuellement prévues ne sont pas consommées. S'investir dans son établissement et élaborer des projets à destination des élèves prend du temps. Moins de postes et plus d'heures supplémentaires, cela signifie aussi moins de dynamisme dans les établissements.

le budget qui leur est consacré n'augmente pas en proportion. Nous notons la volonté de mettre l'accent sur l'école inclusive par la création de 4 000 postes d'AESH, mais nous regrettons qu'il ne soit pas envisagé d'augmenter la rémunération La plupart des AESH sont payés au SMIC en début de carrière et, de fait, il apparaît qu'ils- et surtout elles, car ce sont majoritairement des femmes -sont à temps partiel. Leurs revenus sont donc trop faibles. Leur mission essentielle mériterait d'être revalorisée. Enfin, cette mission englobe l'enseignement agricole, qui est un vrai atout français même si nous en parlons trop peu. Heureusement, je sais que dans cet hémicycle- les orateurs avant moi l'ont dit -nous y sommes toutes et tous très attachés. Son rôle dans la mise en oeuvre de la transition écologique est central, car il est indispensable si nous voulons réussir à inventer un nouveau modèle agricole viable tout en accompagnant et en soutenant pleinement nos agricultrices et nos agriculteurs. Comme pour de nombreux sujets, c'est grâce à l'école que les grandes batailles se gagnent. Ne ratons pas le coche De plus, la décennie à venir connaîtra un grand nombre de départs à la retraite dans le monde agricole. Nous devons être en mesure de préparer la relève. Nous ne pourrons pas relever ces défis sans un enseignement agricole de qualité. Aujourd'hui, cette qualité existe, notamment grâce aux créations de postes intervenues entre 2012 et 2017. Il faut la préserver. Ce budget prévoit la suppression de 80 postes, qui, cumulée aux suppressions précédentes et à venir, porte le total à 300 postes de moins durant votre mandat. En proportion, c'est comme si on supprimait 10 000 postes dans l'éducation nationale : c'est colossal Et l'on nous signale déjà des difficultés pour dédoubler les classes lors des travaux pratiques (TP), pour appliquer les différentes réformes et pour parvenir à l'équilibre des budgets des établissements. Si nous ne changeons pas de cap, nous risquons d'atteindre le point de non-retour. J'espère que, lors de nos débats, nous saurons faire les choix nécessaires pour préserver la qualité de l'enseignement agricole. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons relu ensemble la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. Il leur indiquait notamment ceci : « Je sais quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d'années et ils ne sont point toujours assidus, surtout à la campagne. Ils oublient l'été le peu qu'ils ont appris l'hiver. Ils font souvent, au sortir de l'école, des rechutes profondes d'ignorance et de paresse d'esprit, et je plaindrais ceux d'entre vous qui ont pour l'éducation des enfants du peuple une grande ambition, si cette grande ambition ne supposait un grand courage. Du courage, les personnels de l'éducation nationale n'en manquent pas ! De la patience, de l'écoute, de la passion et de l'innovation, ils en font preuve chaque jour Ce dont ils manquent, monsieur le ministre, c'est de moyens. Ce budget est-il à la hauteur de leur engagement et de leurs besoins au service de nos enfants ? Pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, la réponse est : non ! La parole

mes chers collègues, la crise du coronavirus a bouleversé notre pays comme elle a bouleversé le monde. Tous nos compatriotes ont été impactés par cette pandémie et par les mesures nécessaires prises pour la combattre. Au sein de nos territoires, les fabriques d'avenir que sont nos écoles ont été particulièrement affectées. Je tiens à saluer l'engagement et le dévouement de nos enseignants. Dans des circonstances difficiles, dans un contexte de grande incertitude, ils ont dû agir au jour le jour pour continuer d'accomplir leur mission. Je les Nous avons mesuré lors du premier confinement à quel point la technologie numérique était essentielle à la poursuite de l'activité scolaire, mais aussi au maintien du lien social que l'école permet. Les professeurs et les équipes ont déployé des trésors d'inventivité pour maintenir leur enseignement. Pandémie ou non, le numérique est très utile au fonctionnement des établissements. Il est à ce titre indispensable de continuer la numérisation de l'école et d'y veiller particulièrement au primaire. Comme chaque année, l'enseignement scolaire est la mission la plus importante du budget général et ses crédits sont en hausse. Cela témoigne de la place accordée par notre pays à l'enseignement. L'école de la République joue un rôle essentiel dans notre société, celui d'instruire les plus jeunes de nos concitoyens et de les amener à développer un esprit critique. Samuel Paty y participait avec passion. souhaitons lui rendre hommage, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui sont pleinement engagés au service de l'éducation nationale. Les dépenses de personnel augmentent cette année, bien que le pic démographique ait été atteint en 2016. Depuis cette date, les évolutions démographiques de la population française conduisent à une diminution du nombre d'élèves d'année en année. Si la dépense publique doit être maîtrisée et adaptée au plus près des besoins des Français, cette augmentation de personnel nous paraît toutefois nécessaire. Certes, le nombre d'élèves diminue, mais leur niveau aussi. L'ancien professeur de mathématiques que je suis est très inquiet de l'évolution de la situation. Le niveau des élèves français est en train de décliner. Particulièrement dans ce que fut ma matière, mais également en français, les performances de nos élèves sont à la baisse. Nous devons réagir vite car nous savons que, dans le parcours de l'enfant, les premières lacunes ont tendance à en entraîner d'autres. Nous soutenons l'effort porté sur le primaire. C'est en effet lors de cette étape clé que beaucoup se joue. La réduction démographique devrait avoir des conséquences positives sur les performances des élèves, en réduisant leur nombre par classe. Il ne faut cependant pas compter uniquement sur cette dynamique, car le nombre d'élèves par classe dans le premier degré en France reste actuellement le plus élevé de l'Union européenne. Pour améliorer l'enseignement, l'évaluation est incontournable. Il nous faut identifier les bonnes pratiques et les généraliser. L'effort consenti par la Nation pour l'enseignement scolaire- d'un montant de plus de 55 milliards d'euros -est majeur. Nous devons faire en sorte que chaque euro compte et que l'enseignement dispensé à nos enfants soit de la meilleure qualité. Il ne s'agit pas de mettre en cause le travail de celles et ceux qui se dédient à l'enseignement, mais il nous faut déterminer ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré, identifier les bonnes pratiques et les généraliser. L'année qui s'ouvre verra ce travail d'évaluation poursuivi par le Conseil d'évaluation de l'école. À cet égard, nous souhaiterions, monsieur le ministre, qu'une attention particulière soit portée afin que les langues régionales de France- je pense notamment

Nous devons continuer d'y consacrer les fonds suffisants pour préparer le meilleur avenir possible. Face à la perspective d'une diminution du niveau des élèves, nous devons faire preuve de vigilance et réagir rapidement. Évaluer nos établissements, c'est nous donner la chance d'améliorer notre enseignement. Continuons de viser l'excellence ; notre avenir en dépend. En conclusion, si le groupe Les Indépendants porte un regard bienveillant sur ce budget, je regrette l'insuffisance de considération à l'endroit de l'enseignement agricole privé. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un budget exceptionnel pour l'éducation nationale ; exceptionnel, du fait de la crise sans précédent que traverse notre pays et à laquelle sont confrontés de plein fouet tous les personnels de l'enseignement, de l'encadrement et même de l'entretien. Ils et elles font tous partie de la première ligne. Que ce soit dans l'enseignement primaire ou secondaire, ils et elles ont mis en oeuvre les conditions d'accueil les plus favorables pour tous les élèves, ils et elles ont organisé les classes, se sont convertis en un temps record à l'enseignement « en distanciel repris, ont veillé au respect des gestes barrières et ont dialogué avec les parents inquiets sans compter leurs heures ni leurs efforts. Nous devons aujourd'hui collectivement leur rendre hommage. Au-delà de notre soutien moral, ce dont le personnel de l'éducation a besoin, c'est une aide à la fois financière et matérielle, et un soutien sans réserve de son administration. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui.

des élèves en situation de handicap. Si nous tenons à saluer cet effort sans précédent en faveur de l'école inclusive, nous proposerons toutefois de revaloriser la rémunération des AESH. L'effort global pour l'enseignement scolaire est important, et il doit être salué ; mais est-il suffisant ? Nous n'en sommes pas persuadés. Monsieur le ministre, dans cette crise, écoutons les personnels de l'enseignement et ce qu'ils ont à nous dire. Écoutons le désarroi des directeurs et directrices d'école au bout du rouleau, qui n'en peuvent plus de devoir mettre en oeuvre sans préavis des protocoles sanitaires qui changent parfois au bout de deux jours, qui sont quelquefois contradictoires et toujours mal expliqués. Écoutons la colère des enseignants du secondaire, qui se sont mobilisés le 10 novembre dernier pour appeler à davantage de moyens pour se protéger et protéger leurs élèves du virus dans les classes bondées des collèges, dans les cantines ou dans les couloirs. Écoutons ces mêmes enseignants du secondaire, qui verront 1 800 postes supprimés dans leurs rangs, et à qui on demandera de faire davantage d'heures supplémentaires alors même qu'ils sont au maximum de leurs capacités. Écoutons les AESH, dont 93 % sont des femmes, âgées en moyenne de 45 ans, qui effectuent un travail indispensable d'accompagnement dans plusieurs établissements à la fois et qui ne gagnent en moyenne que 760 euros par mois, soit 300 euros de moins que le seuil de pauvreté. Ce que le corps pédagogique demande est simple et revient dans chacune des prises de parole de ses représentants : plus de personnel, plus de moyens, plus de salaire pour faire leur métier dans les meilleures conditions. Épuisés par la crise, les personnels de l'éducation ne supporteront pas de nouvelles suppressions de postes ni des horaires extensibles comme cela est proposé dans ce PLF. Écoutons-les maintenant et, surtout, agissons pour eux. Enfin, je souhaite attirer votre attention, mes chers collègues, sur les échanges que nous avons eus concernant le rétablissement des valeurs de la République au sein de l'école. Les faits qui ont animé nos débats sont connus de tous des élèves qui boudent, qui trouvent des justifications aux assassins de Samuel Paty ou de, ou encore des vidéos insoutenables de décapitation qui circulent sous le manteau. Mes chers collègues, les enseignants qui dédient leur carrière et parfois leur vie à l'éducation des générations futures font plus que savoir ce que signifient les valeurs de la République : ils et elles les incarnent au quotidien. La République n'est pas une leçon ni un programme scolaire qui doit être remanié pour être mieux appris. C'est une dynamique, un processus toujours en cours, toujours vivant. C'est une marche collective vers l'émancipation, qui se construit ensemble à travers les générations vers un destin commun. Les enseignants et enseignantes ne sont pas les dépositaires d'une vérité absolue que les élèves doivent réciter le petit doigt sur la couture du pantalon : ils sont au contraire les animateurs d'un projet commun. Ils ne sont pas que les gardiens d'un ensemble de règles : ils sont aussi ceux qui partagent et mettent en oeuvre notre idéal collectif. Pour y parvenir, il faut que cet élan se remette en marche, que les enseignants se sentent de nouveau au coeur de notre République, que les moyens soient mis à leur disposition et que le soutien de la société se manifeste par des preuves concrètes, donc financières. C'est par la mise en pratique concrète des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité que la République sera partagée et embrassée par tous, pour qu'ainsi les élèves en soient témoins, qu'ils voient que la République sait se montrer aussi généreuse avec celles et ceux qui la font vivre qu'intransigeante envers ceux qui la combattent. Tel est idéal que nous appelons de nos voeux.

primaire, qui, pendant trop d'années, avait été délaissée, alors que- nous le savons -, faute de moyens suffisants, les inégalités de réussite en fonction de l'origine sociale s'y creusent et s'y sédimentent le plus souvent.

d'étendre le dédoublement des classes aux grandes sections de maternelle en éducation prioritaire, de ne fermer aucune école rurale, sauf en cas d'accord du maire, et d'améliorer les conditions de travail des directeurs d'école. Grâce à l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans, 26 000 élèves supplémentaires sont accueillis depuis la rentrée 2019 en maternelle. Des crédits de 100 millions d'euros sont ouverts pour accompagner les communes à ce titre. cette mesure est venue autant traduire un engagement de campagne que satisfaire les revendications exprimées par d'autres responsables politiques avant 2017, mais non traduites dans les faits.

pour les communes qui souhaitent conserver la semaine de plus de quatre jours. L'augmentation des crédits pour le second degré se traduira par un volume d'heures supplémentaires de près de 1 000 équivalents temps plein. Ce budget engage la revalorisation du métier d'enseignant et le renforcement de l'attractivité des métiers de l'éducation. En attendant les conclusions du Grenelle de l'éducation, une revalorisation de 400 millions d'euros est d'ores et déjà inscrite au budget, de même que la création d'une prime d'équipement informatique de 150 euros net. net. Visant le même objectif, d'autres politiques soutenues par ce budget doivent être citées : je pense aux 3 000 étudiants supplémentaires qui auront accès à une préprofessionnalisation de trois ans à partir de la deuxième année de licence ; je pense également aux élèves inscrits en master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, qui pourront désormais être accueillis en stage en alternance pendant leur deuxième année de master. Nous resterons attentifs à la reconnaissance de ces métiers essentiels. François Dubet et Marie Duru-Bellat rappelaient dans un ouvrage récent que les vaincus ont vu leur situation se dégrader ces dernières décennies, que l'on retrouve dans la vie politique elle-même entre les élites éclairées et instruites et tous ceux qui se sentent dépossédés et méprisés. C'est le sens de ce budget comme des précédents que de répondre à ce constat. Alors que la crise du covid-19 risque de produire des effets négatifs cumulatifs,

Ce sera aussi l'objet du Grenelle de l'éducation et de la refonte de la carte REP+ sous la forme d'une expérimentation annoncée dimanche dernier. Des préconisations renforcées pourraient être faites au service d'une politique plus fine, permettant l'indexation des moyens en fonction d'un indice de mixité sociale.

la mission « Enseignement scolaire » prend cette année un relief particulier en raison de la pandémie qui a bouleversé l'organisation des cours. À cette difficulté s'est ajouté l'impensable : le tragique assassinat du professeur Samuel Paty ; un acte odieux, attaquant la République en général et la liberté d'enseigner en particulier. Avec 76 milliards d'euros demandés pour 2021, il est coutume de dire que l'enseignement scolaire est le premier poste de dépenses au sein du budget général. Aussi, nous attendons beaucoup de notre système d'éducation nationale. Faut-il rappeler que l'école est le ciment de notre pacte républicain ?

Il est en effet fondamental de persévérer dans la réduction des inégalités sociales. L'absence d'égalité dans les conditions d'apprentissage est la garantie d'une reproduction permanente des inégalités de destin. que le budget de la mission traduit une volonté de renforcer, en 2021, les moyens de l'éducation nationale. Alors que le nombre d'élèves diminue, les crédits de paiement ainsi que les autorisations d'engagement augmentent d'un peu plus de 2 % ; nos collègues rapporteurs l'ont souligné. C'est une équation positive, bien que je regrette un schéma d'emploi défavorable au secondaire, alors que les classes y sont également trop chargées. Je souligne que le décrochage scolaire lié à la pandémie concerne d'abord les jeunes des lycées d'enseignement professionnel. Il faudra prévoir un plan de rattrapage pour ces établissements. N'oublions pas qu'on y forme nombre de ceux qui étaient en première ligne pendant la crise sanitaire.

En revanche, je souhaite souligner les efforts qui sont portés en faveur des enfants en situation de handicap. L'école n'est toujours pas suffisamment inclusive. le recrutement de 4 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap va dans le bon sens, nous partons de loin : il faudra donc faire plus pour une école accessible à tous. En écho à une autre politique de votre gouvernement, monsieur le ministre, il faut « 1 élève 1 solution

Malgré la mobilisation extraordinaire du corps enseignant, la crise sanitaire a délégué une partie de l'instruction à la famille, avec toutes les inégalités sociales que l'on imagine. J'y ajouterais la question de l'accès au numérique. Dans le contexte du recours à l'enseignement à distance, la fracture numérique nous est apparue encore plus cruelle pour les familles des territoires ruraux. vous n'ayez pas la tutelle du secteur numérique, permettez-moi d'en appeler, sur ce sujet, à la responsabilité du Gouvernement. Je citerai une phrase de notre regretté collègue Alain Bertrand, extraite de son rapport sur l'hyper-ruralité Finalement, en ne construisant pas un modèle économique de desserte numérique et de téléphonie mobile à l'échelle du territoire national, l'État a organisé dès l'origine un système de creusement de l'inégalité territoriale d'accès à des services pourtant pourtant devenus universels et d'autant plus stratégiques dans les zones de faible densité. » C'est un fait. Plus favorable aux territoires, la dotation de 50 millions d'euros pour soutenir la réhabilitation par les collectivités locales des bâtiments d'internat ainsi que la poursuite du plan Bibliothèques, qui bénéficie aux zones rurales, méritent d'être soulignées.

Mais l'école, ce sont aussi des professeurs, et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'école de la confiance sans professeurs en confiance. Permettez donc au professeur que je reste de rappeler dans cet hémicycle la réalité de ce que vivent les enseignants, réalité, qui, je le crois, nous aidera à comprendre l'urgence de renouer un pacte de confiance entre les professeurs, l'école et la société. Je ne peux m'empêcher ce matin, en évoquant des professeurs, de penser à Samuel Paty. Il s'inscrivait dans une longue lignée, nous rappelant que notre école fut fondée pour partie par des professeurs, au point que l'on a pu parler, voilà cent ans, de « la République des professeurs », âge d'or mythifié durant lequel ils auraient bénéficié d'un prestige et d'une autorité incontestée. Ce temps, bien sûr, n'a jamais existé. Les maîtres ont toujours eu des raisons de se plaindre de leur condition au sein de la société. Aujourd'hui, les craintes d'entrer dans la carrière, le découragement des plus jeunes expédiés comme des Marie-Louise dans les territoires les plus difficiles, la lassitude des plus chevronnés, témoignent de la perte d'attractivité d'un métier exceptionnel. Des signes d'espérance apparaissent. Le professeur que l'on pensait condamné par l'ordinateur retrouve sa place et l'école à distance nous rappelle ce que disait déjà Jules Ferry en 1879 : « Celui qui est maître du livre est maître de l'éducation. Enseigner est un métier exigeant qui nécessite appétence, compétences et formation. Voilà ce que de nombreux parents ont découvert, ou redécouvert, lors du premier confinement.

Monsieur le ministre, ce pacte de confiance nécessite à l'évidence un rattrapage en termes de rémunérations, de conditions de travail, d'humanisation et d'individualisation des carrières. Le Grenelle de l'éducation doit apporter des réponses précises à ces questions. Les tensions apparues cette semaine et les claquages de portes enregistrés voilà trois jours ne nous rassurent pas. Certes, la hausse des crédits, notamment ceux qui sont affectés à la revalorisation des traitements, la création d'une dotation d'équipement informatique, l'instauration d'une prime d'attractivité de début de carrière, sont de bonnes mesures. Cependant, l'effort devra être mené dans la durée et ne pourra pas se cantonner à des avancées matérielles. Comme les hussards noirs de la III République, les professeurs du XXI siècle doivent être armés philosophiquement pour combattre ceux qui veulent abattre la République.

La formation continue des professeurs sera-t-elle érigée en impérieuse nécessité par un ministère qui la considère depuis si longtemps comme une variable d'ajustement ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous constatons de manière factuelle une hausse substantielle du premier budget de l'État,

S'il ne fallait retenir qu'un seul marqueur de ce budget, je citerais l'effort à destination du service public de l'école inclusive, qui est désormais doté d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Je connais trop la détresse des familles qui ne peuvent pas scolariser leur enfant par manque d'un accompagnement à l'école pour ne pas insister sur cette action.

Toutefois, au-delà de ce satisfecit quantitatif, la revalorisation salariale de ce métier me semble absolument indispensable. Je partage également la conviction qu'il faut

alors que la Cour des comptes persiste à pointer l'inefficacité de l'éducation prioritaire sous sa forme actuelle. L'annonce discrète d'une expérimentation qui pourrait préfigurer une prochaine réforme montre bien la délicatesse d'un chantier que l'exécutif prend soin de reporter au-delà de 2023.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec humilité et émotion que j'interviens pour la première fois à la tribune du Sénat, comme nouveau sénateur de Saône-et-Loire.

de poursuivre des études supérieures. De nombreux projets post-bac sont ainsi bloqués, faute de moyens. Bien plus, ce budget n'est pas à la hauteur de l'ambition agricole qui devrait être celle de notre pays. La France doit soutenir la nouvelle génération d'agriculteurs dans sa volonté d'innover, de faire évoluer les productions et de prendre en compte les enjeux environnementaux. C'est pourquoi le programme 143 devra être beaucoup plus ambitieux.

Prenons garde, monsieur le ministre, que la broyeuse de Bercy ne vienne faucher le blé encore vert et n'ensevelisse dans son sillon les espoirs de l'enseignement agricole, n'enterre la vocation agricole de notre pays et n'enfouisse pour longtemps l'espérance de voir notre agriculture relever les défis du futur. C'est alors toute la société qui y perdrait. La parole

Le budget de la mission « Enseignement scolaire » pour 2021 s'établit à 53,6 milliards d'euros, hors cotisations aux pensions de l'État, soit une augmentation de plus de 3 %, avec 1,6 milliard d'euros supplémentaires.

Marie-Pierre Monier. Cet amendement vise à financer la titularisation d'une partie des contractuels de l'enseignement secondaire. Alors que le Gouvernement réduit les effectifs dans le second degré, il est proposé de titulariser chaque année 10 % des agents contractuels, sous condition d'ancienneté. Le nombre des contractuels, qui atteint 40 % dans certaines zones tendues où le recrutement d'enseignants reste difficile dans certaines matières, est en contradiction avec l'exigence de stabilité des équipes, élément pourtant déterminant d'une politique tournée vers la réussite des élèves. L'éducation nationale a aujourd'hui régulièrement recours aux enseignants non titulaires, qui sont environ 37 000. Ces postes précaires mettent les enseignants dans des situations difficiles, instables, qui ne favorisent ni leur épanouissement personnel ni le bon exercice de leur métier. En effet, ils doivent s'adapter, sur des périodes très courtes,

Ces enseignants ont, pour certains, de nombreuses années d'expérience. Ils doivent pouvoir être titularisés en fonction de la qualité de leur enseignement et des critères validés par le dialogue social au sein de l'institution, sans avoir à réussir les concours internes. Malgré le plan institué par la loi Sauvadet en 2012, le processus de titularisation fonctionne mal. Pourtant, la qualité du travail fourni par les contractuels nécessiterait une reconnaissance et une intégration dans les corps de l'État. Il serait nécessaire de mettre en place un nouveau dispositif qui prenne la suite, tout en l'améliorant, et qui tienne compte de l'expérience de ces contractuels.

En revanche, les conditions de rémunération de ces personnels doivent également faire l'objet de notre attention. En effet, 72 % des AESH sont rémunérés à l'indice plancher de leur grille de salaire ; en moyenne, un AESH gagne 760 760 euros par mois. Pour rappel, le seuil de pauvreté relative, qui correspond à 60 % du revenu médian, s'établit à 1 063 euros par mois, et le seuil de pauvreté monétaire qui est fixé, lui, à 50 % du revenu médian s'élève à 885 euros par mois. Dans les deux cas, les AESH en sont très loin. De plus, bien souvent, au vu du nombre d'heures effectuées et des déplacements qu'ils sont obligés de réaliser, les AESH n'ont pas l'occasion de prendre un deuxième travail pour augmenter un peu leurs revenus. Monsieur le ministre, voilà une catégorie de personnels dévoués qui mériteraient un peu plus de la part de l'État. C'est pourquoi nous proposons de poser, dès ce projet de loi de finances, un premier acte fort : ce serait un signal pour montrer aux AESH qu'ils ne sont pas oubliés. Nous proposons d'augmenter de 10 % l'enveloppe globale allouée personnels pour porter leur rémunération moyenne à 836 euros, ce qui les rapprocherait au moins du seuil de pauvreté monétaire. C'est loin d'être suffisant, mais nous appelons aussi le Gouvernement à nous emboîter le pas pour abonder cette enveloppe au-delà de ce que les règles de la discussion budgétaire nous autorisent à

dès lors qu'il y a là un véritable sujet. Cette indemnité constituerait donc une amélioration significative de leurs conditions salariales : ce sont 20 millions d'euros qu'il faudrait pour l'exercice 2021.

du Gouvernement ? La situation des AESH mérite évidemment le débat que nous avons et l'intérêt que vous manifestez.

débouchent sur des CDI, ce dont nous sommes fiers et heureux, car c'est bon pour tout le monde. Nous sommes aussi en train de travailler à la fluidité des carrières. Nous avons ainsi créé des AESH référents, qui perçoivent une indemnité annuelle leur permettant d'améliorer un peu leur pouvoir d'achat.

et que les PIAL étaient une sorte de machination infernale, là où il y a au contraire le début d'une politique cohérente. Il faut reconnaître, même s'il reste du chemin à parcourir, que jamais autant n'a été fait pour l'école inclusive.

Il n'y a pas grand-chose qui puisse justifier une telle mesure. Je ne reviens pas sur les questions salariales. Devoir enchaîner plusieurs postes, y compris en ville-

de vote. J'insiste sur le nécessaire accompagnement des élèves les plus en difficulté vers la réussite. En tant qu'ancienne adjointe aux écoles et maman d'un enfant en situation de handicap, je mesure pleinement l'engagement de ces personnels et les difficultés qu'ils rencontrent, mais également les améliorations dont ils bénéficient

trop faibles empêchent certains établissements, notamment les plus petits, situés en zone rurale, de proposer certaines matières. Que l'on partage ou non l'esprit de cette réforme sur le fond, il n'en reste pas moins que son objet était de permettre aux élèves de sortir des logiques de filières et de choisir parmi un plus large panel de matières. Or, dans les faits, ce n'est possible que dans certains grands établissements. L'augmentation du nombre de postes pourrait favoriser l'augmentation de la DGH dans de nombreux petits établissements d'enseignement secondaire,

La loi d'orientation des mobilités de 2019 prévoit un programme d'apprentissage du vélo pour tous, afin de permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public. Nous nous réjouissons naturellement de cette mesure, puisque l'école est le bon vecteur pour diffuser au sein de la société la pratique du vélo, moyen de transport quotidien parmi les moins polluants et extrêmement positif en termes de santé et de pratique physique.

Mes chers collègues, au lieu de vous présenter un énième amendement d'appel, nous vous proposons de voter, dès ce projet de loi de finances, les crédits du « Savoir rouler à vélo ». Nous proposons ainsi de doter chacune des 50 130 écoles que compte notre pays de 1 000 euros, soit une enveloppe de 50,13 millions d'euros, afin de leur permettre d'acheter des vélos et de former les personnels.

en toute sécurité, car nous constatons l'émergence d'une véritable « génération vélo ». L'objectif est de permettre aux élèves de maîtriser la pratique du vélo au moment de leur entrée au collège, comme le précise la loi. Celle-ci indique également que « cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire ». Nous avons bien conscience que le dispositif dépend avant tout des moyens de la jeunesse et du sport. Toutefois, les écoles étant formellement visées par la loi, nous souhaitons savoir comment elles seront dotées, ainsi que les communes qui seraient susceptibles d'être mises à contribution.

maturité. Le temps scolaire est un temps limité. Au détriment de quels enseignements le vélo serait-il enseigné ? Par quels moyens et avec quelles compétences ? J'ajoute que, heureusement, les parents-

offerte de revenir à l'un de mes marronniers favoris. Chaque fois qu'un débat de cette nature a lieu dans cet hémicycle, je reviens à la charge

le sport ! En plus d'être un savoir fondamental, il est aussi déterminant pour la santé, l'agilité, la vélocité, etc. : autant de qualités indispensables dans le monde d'aujourd'hui.

Pas besoin d'en faire une guerre de religion

que l'on doit notamment à la possibilité d'avoir des effectifs réduits, de dédoubler les classes, chaque fois que c'est nécessaire pour l'organisation de travaux pratiques en toute sécurité. Cela implique donc de disposer suffisamment de postes d'enseignants.

tous les dédoublements nécessaires, ce qui oblige certains établissements à renoncer à l'organisation de certains travaux pratiques- on m'a cité l'exemple du travail avec les grands animaux -pour des motifs de sécurité des élèves. De plus, le manque de postes associé à la mise en place de la réforme du lycée dans les lycées agricoles crée quelques situations ubuesques.

Pourtant, l'enseignement agricole est amené à relever de nombreux défis. Il faut attirer de nouveaux élèves puisque, je le rappelle, la moitié des agriculteurs partiront à la retraite d'ici dix ans.

professionnels. Selon l'exposé des motifs, il s'agit de financer des recrutements d'assistants d'éducation « afin de permettre aux enseignants vulnérables de dispenser leurs cours à distance tout en maintenant un encadrement des élèves dans les établissements

du lycée Henri-Queuille de Neuvic, sur le plateau de Millevaches, qui continue à aider les agriculteurs à développer des filières d'excellence.

cette affaire pour que, une fois que vous aurez levé le gage, le Gouvernement soit enfin cohérent

d'euros. La réussite de tous les élèves implique de doter les enseignants d'une formation initiale et continue de qualité tout au long de leur carrière. Pourtant, ces derniers nous font souvent part de leur insatisfaction à ce sujet, due à l'offre restreinte qui leur est proposée. Il est essentiel que la formation des enseignants permette un approfondissement sérieux des contenus didactiques. Elle doit s'inscrire dans une approche « sur demande », au plus près de leurs attentes et de leurs besoins, qu'ils soient liés à leurs disciplines ou à leurs aspirations personnelles. Le schéma directeur de la formation continue des personnels de l'éducation nationale doit évoluer en conséquence, dans une logique de concertation avec les équipes.

Ces fonds sont versés aux établissements pour apporter une aide exceptionnelle aux familles défavorisées qui en ont le plus besoin. Leur but est de compléter les dispositifs correctifs des inégalités sociales et matérielles des familles, afin que la réussite de tous les élèves puisse être au rendez-vous.

peinent à assumer leurs missions de lutte contre les difficultés scolaires. Les besoins en postes existaient avant la crise sanitaire ; ils n'ont pas disparu depuis. C'est pourquoi un moratoire sur la fermeture des postes en Rased devrait être appliqué. Il faut également dresser une carte des renforts nécessaires en lien avec le collectif national

tous les temps périscolaires de garderie et de cantine. En effet, si les AESH interviennent principalement dans le temps scolaire, ils peuvent être notifiés pour des activités périscolaires, comme la

vise à augmenter les moyens consacrés aux lycées professionnels. La réforme de l'enseignement professionnel avait pour objectif de faire de la voie professionnelle un parcours de réussite et d'excellence pour ses élèves : aussi,

constate des transferts de la voie professionnelle vers les voies technologique et générale, ainsi que des réductions d'horaires dans certaines disciplines. Dans ce contexte, les lycées professionnels seront peu en mesure de prendre en compte les évolutions et les transitions nécessaires sur le marché de l'emploi pour leurs élèves.

des élèves de lycée professionnel. Je rappelle que, à la rentrée, on recensait 2 574 emplois d'enseignants du second degré public exerçant la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.

Plus que jamais, nous devons permettre aux établissements à rythme approprié, notamment les maisons familiales rurales (MFR), de continuer à rayonner sur le territoire national- et au-delà, d'ailleurs. Nous en avons tous dans nos départements et nous connaissons leur excellence. Ces établissements participent à l'animation des territoires ruraux, voire très ruraux, leur taux d'insertion professionnelle est remarquable et, à ce jour, inégalé. Ils savent aller chercher des jeunes aux profils toujours singuliers, dont certains sont en difficulté, voire en échec, dans l'institution scolaire classique, pour les amener, par une autre pédagogie, à la réussite professionnelle. Ils auraient toute leur place dans le dispositif « 1 jeune, 1 solution » mis en place par le Gouvernement. Pourtant, aucune mesure spécifique les concernant n'est prévue. J'ai visité cette semaine la MFR de Vayres, dans mon département. J'y ai trouvé un précipité d'audace et une ambiance de travail que nombre d'établissements envieraient. de leur statut associatif unique, de leur créativité et des liens forts qui se nouent entre les formateurs, les jeunes et leurs familles, les MFR sont une bouffée d'oxygène dans un monde si morose. Quand j'ai interrogé Victor, Camille, Chloé et les autres sur la façon dont ils voyaient les choses, j'ai été saisie par leurs réponses : ces jeunes croient en l'avenir, en leur projet. Ils ont tous des parcours multiples, riches de diverses expériences acquises en alternance. Ils croient en leur territoire, en leur terroir, qu'ils aiment. Pourtant, ce projet de loi de finances ne leur rend pas hommage. Le coût unitaire de formation par élève versé par l'État est en moyenne de 9 900 euros pour les établissements agricoles publics,

par manque de moyens. Il me semble absolument essentiel de développer cet outil. Monsieur le ministre, j'ai un peu de mal à comprendre votre position depuis le départ. Je vous ai entendu, Étang-sur-Arroux, dans mon département, en présence du Président de la République, exprimer votre attachement, votre amour même, pour l'enseignement agricole. Vous avez ensuite accueilli les élèves de Saône-et-Loire

les chiffres de mortalité par noyade sont en progression constante et il est urgent que l'ensemble des jeunes de notre pays sachent nager. Aujourd'hui, on estime que 50 % des enfants ne possèdent pas cette

nationale. C'est particulièrement vrai dans le second degré, dans le cadre de l'éducation physique et sportive, mais nos efforts vont tout particulièrement porter sur le premier degré. C'est la raison pour laquelle on parle d'aisance aquatique avant même de parler de savoir nager. Ces actions vont beaucoup concerner la coopération entre le monde associatif

Le Gouvernement annonce la création de 250 ULIS en lycée sur le quinquennat. Il faut un investissement similaire dès le premier degré pour permettre la création de dispositifs d'accompagnement adaptés à tous les élèves. cet amendement permettrait notamment d'augmenter le nombre de classes ULIS dans les territoires ruraux dans lesquels, bien trop souvent, les élèves de ces classes doivent parcourir de très longues distances pour aller à l'école, ce qui complique encore davantage leur scolarité.

de la rémunération des médecins de l'éducation nationale. » Il propose une revalorisation indemnitaire de 30 % afin de se rapprocher du niveau de rémunération des médecins inspecteurs de santé publique. Le coût de cette mesure est estimé à 3 millions d'euros. Cette revalorisation est indispensable, alors que de nombreux postes de médecins scolaires sont vacants

les écrans ont envahi la vie des enfants ; on poursuit la fuite en avant sans débat sur la 5G. Tout cela conduit à la sédentarité, à l'obésité et à la maladie. D'un côté, on essaye de réparer, mais, de l'autre, on casse.

L'amélioration des conditions d'exercice des directeurs d'école est l'un des principaux chantiers que nous menons, vous le savez. En cette fin de mois de novembre, la prime de 450 euros que nous avons mise en place est versée. Une série de

dans les obligations de service des professeurs du premier degré. Nous avons également affecté 12 500 jeunes du service civique en appui aux directeurs. Enfin, une fonction de directeur référent auprès des directeurs académiques est en train d'être expérimentée. Une enveloppe de 21 millions d'euros sera consacrée à une augmentation pérenne des directeurs d'école l'an prochain, qui s'ajoute à ce que nous avons fait cette année, avec cette prime de 450 euros par directeur. Enfin, le Grenelle de l'éducation a mis cette question en son centre.

Assemblée, pour la bonne raison que l'enseignement agricole repose très largement sur l'internat et que les relations entre les enseignants, les élèves et les moniteurs y sont de nature assez différente.

certains établissements, faute de personnel en nombre suffisant. Or il importe que ces trois séances annuelles d'éducation à la sexualité puissent avoir lieu, car elles constituent un outil indispensable à la déconstruction des stéréotypes de genre, à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la prévention contre les pratiques sexuelles à risque des jeunes.